contre 21 % dans les autres familles. La pension alimentaire, qui vise à couvrir partiellement les dépenses liées à l’entretien et à l’éducation des enfants, est aujourd’hui considérée comme un revenu imposable. Cela aboutit à une double peine pour les parents seuls, majoritairement les mères, comme je Non seulement elles paient plus d’impôts, mais elles voient leurs droits sociaux diminuer, ceux ci étant souvent soumis à des conditions de ressources. Il est donc essentiel de corriger cette anomalie fiscale, afin de mieux protéger ces familles vulnérables et réduire les inégalités socioéconomiques.

tout en limitant les effets de déductibilité asymétriques.

Hochart. Le présent amendement vise à encadrer l’avantage fiscal lié à la déduction des pensions alimentaires, en réservant celle ci spécifiquement aux parents résidant en France. Actuellement, les pensions alimentaires versées à des proches, comme les parents, sont déductibles des impôts sous certaines conditions, indépendamment du lieu de résidence du bénéficiaire. Ainsi, nous proposons de restreindre cet avantage aux pensions versées aux parents résidant sur le territoire national. Le motif économique Tout d’abord, il s’agit de garantir que les contribuables bénéficiant de cet allégement fiscal contribuent directement à l’économie et au système fiscal français. Ainsi, nous nous assurons que les fonds restent dans le circuit économique national, ce qui est essentiel pour financer les services publics et maintenir la solidarité nationale. de cet amendement répondent à une préoccupation croissante concernant le risque d’évasion et de fraude fiscales, lié aux versements effectués à des bénéficiaires vivant à l’étranger. En effet, il est souvent difficile de contrôler l’utilisation des fonds versés hors de France ou de vérifier la légitimité des pensions alimentaires. Dans ces cas, en restreignant l’avantage fiscal aux seuls résidents français, nous réduisons les risques d’abus et de détournement

père survenu en 2011. Alors que des efforts significatifs sont demandés aux contribuables français, il est temps d’agir de manière plus efficace contre la fraude. L’adoption de cet amendement permettrait non seulement de mieux protéger nos finances publiques, mais aussi de redonner du sens à l’équité fiscale et à la confiance dans le système. Quel est l’avis de la commission ? En prétendant

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Depuis une loi adoptée en 2000, le régime fiscal de la prestation compensatoire prévoit que, si le capital est libéré en numéraire sur une période supérieure à douze mois à compter de la date du jugement, le débiteur – l’homme, en

deuxièmement, l’exonération partielle des indemnités temporaires servies aux victimes d’accidents du travail ; troisièmement, l’exonération des prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles

Je comprends l’objectif de simplification et de réduction du nombre des dépenses fiscales, mais la suppression sèche de ces trois dispositifs, qui n’ont pas été évalués depuis 2011, me paraît, à ce stade, disproportionnée.

je rappelle que les indemnités temporaires ne sont exonérées qu’à hauteur de 50 % de leur montant. Seules les prestations et les rentes viagères sont totalement exonérées.

l’avis du Gouvernement ?

les seuls salariés et remettraient donc en cause des évolutions législatives récentes qui tendent à aligner le traitement fiscal des salariés et des non salariés placés dans la même situation.

Face à une augmentation du coût de la vie, marquée notamment par l’explosion des prix de l’énergie et des produits de consommation courante, il est impératif de garantir une égalité fiscale entre l’ensemble des professions. Alors que de nombreux Français peinent à boucler leurs fins de mois, le maintien d’un tel avantage pour les journalistes, hérité d’une autre époque, ne peut plus être justifié. Cette suppression s’inscrirait dans une démarche de rationalisation des dépenses fiscales, doivent être réservées à des objectifs stratégiques ou sociaux clairement identifiés, dans un souci d’équité. Il est indispensable de mettre fin à des dispositifs qui créent des inégalités et alimentent un sentiment d’injustice parmi les contribuables. La situation budgétaire de la France nécessite de repenser l’ensemble des niches fiscales, afin de ne conserver que celles qui répondent à un intérêt général

de dégagisme. Une démocratie repose sur des élus qui s’engagent. Il est normal qu’ils perçoivent une indemnité de fonction, quel que soit leur niveau de responsabilité et quelle que soit l’assemblée dans laquelle ils siègent, puisqu’ils ont ainsi acquis une légitimité.

du précédent, cet amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi si celui ci est annulé et que le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise. En fait, il s’agit d’un alignement sur les conditions fiscales qui s’appliquent aux indemnités de licenciement sans cause réelle

Quel est l’avis de la commission ?

L’article 7 de la loi de finances pour 2024 prévoit également une majoration pérenne de 100 euros des plafonds d’exonération fiscale pour la « prime transport », la portant

afin de pallier la pénurie croissante de praticiens dans certaines régions. Le système de cumul emploi retraite a permis à de nombreux médecins et infirmiers retraités de poursuivre leur activité, contribuant ainsi à la prise en charge des patients, en particulier dans les zones rurales rurales ou sous médicalisées. En exonérant ces revenus d’impôt, nous cherchons à rendre le cumul emploi retraite plus attractif et à renforcer l’offre de soins dans les territoires où les déserts médicaux se font de plus en plus prégnants. Cette réforme vise à soutenir notre système de santé en facilitant la réintégration de ces professionnels,

Il s’agit par ailleurs d’une mesure pérenne et juste, qui permettrait notamment d’éviter la suppression massive des allégements de charges sur le travail.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

Aujourd’hui, chacun des deux premiers enfants permet de bénéficier d’une demi part fiscale. Ce dispositif n’est plus en adéquation avec la situation du pays. Cet amendement vise donc à accorder une part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Son adoption permettrait à la fois de soutenir une politique de natalité et de rendre du pouvoir d’achat

j’ai cru comprendre que, comme nous, vous souhaitiez que les comptes publics soient bien tenus. Or vous proposez une mesure

à M. Bernard Delcros. Le contrat d’épargne handicap est un produit d’épargne qu’une personne en situation de handicap souscrit pour se garantir le versement de revenus futurs.

je vous propose de le faire évoluer pour le porter à 1 616 euros, soit une majoration de seulement 91 euros par an et de moins de 8 euros par mois. Le montant de cette majoration est certes très limité, mais sa portée concrète et symbolique serait réelle pour nos concitoyens en situation de handicap.

modestes. Monsieur le ministre, vous m’objecterez sans doute qu’il faudrait plutôt envisager une réforme structurelle de la branche autonomie pour financer plus durablement les frais de dépendance et d’hébergement des personnes âgées dépendantes.

concrète et immédiate, sans pour autant fermer la porte à une réflexion plus structurelle. L’amendement

et accueillies dans un Ehpad ou dans un établissement de soins de longue durée bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée. L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables, excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie, à revenu modeste, hébergées en établissement. À domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent, quant à elles, bénéficier d’un crédit d’impôt, et cela depuis 2017. Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit lorsqu’elle entre en établissement, à la suite d’un accident de la vie ou de l’apparition de troubles du comportement sévères. On évalue à au moins à au moins 25 000 euros par an les frais de séjour en établissement spécialisé, de sorte que les familles doivent être mises à contribution.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

tout à fait favorable

Dans ce système, les résidents les plus aisés sont notoirement mieux aidés que ceux qui disposent de moins de ressources. À l’inverse, 76 % des résidents ne peuvent pas couvrir financièrement leurs frais de séjour avec leur revenu courant. Voilà une injustice fiscale particulièrement insoutenable à l’heure où le sujet du pouvoir d’achat des petites retraites est brûlant et où la réforme du modèle des Ehpad reste au milieu du gué. Dans ce contexte, cet amendement de notre collègue Éric Gold vise à introduire une mesure qui fait largement consensus.

Il pourrait donc être intéressant d’utiliser ce PLF pour introduire des mesures concrètes de justice sociale en faveur des résidents d’Ehpad les plus modestes. La parole

nous transformions la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissements spécialisés en un crédit d’impôt. Le coût de cette dépense fiscale est estimé, pour 2023, à près de 272 millions d’euros d’euros pour plus de 424 000 bénéficiaires. La réduction d’impôt s’élève à 25 % des dépenses engagées au titre de la dépense et de l’hébergement des seules personnes dépendantes hébergées dans un établissement spécialisé, à l’exclusion des dépenses de soins, qui sont couvertes par la sécurité sociale. le dispositif sont plafonnées à 10 000 euros par an et par bénéficiaire. Par ailleurs, cette réduction d’impôt est cumulable avec le bénéfice d’autres aides, qui prennent en charge tout ou partie des frais associés à l’hébergement des personnes. Dans le rapport que Christine Pirès Beaune a remis à la Première ministre en juin 2023, notre collègue considère que la transformation en crédit d’impôt de ce dispositif fiscal le rendrait plus redistributif. En effet, si le montant total des restes à charge est plus élevé pour les bénéficiaires de la réduction d’impôt, il représente néanmoins une part moins importante de leurs ressources, le taux d’effort passant à 90 % contre 150 % aujourd’hui.

que nous transformions la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissements spécialisés en un crédit d’impôt.

Or, si la réduction d’impôt est plafonnée à 10 000 euros, le montant médian des aides sociales à l’accueil par bénéficiaire s’élève à 4 900 euros par an. En outre, la réduction d’impôt est cumulable avec les aides sociales départementales. Le montant de la prise en charge des départements est donc infime

Nous suivons en cela la préconisation de la Cour des comptes figurant dans le rapport de mars 2024 sur le soutien de l’État aux services à la personne, qui conseillait de restreindre ce crédit d’impôt aux activités de la vie quotidienne et de réallouer une partie de son produit aux branches famille et vieillesse de la sécurité sociale.

qui constitue, semble t il, la deuxième dépense fiscale la plus importante pour les finances publiques. Le coût de ce dispositif, qui profite à l’ensemble des contribuables, est en constante augmentation : il s’est élevé à 6 milliards d’euros en 2023 pour 4,7 millions de foyers, soit une hausse de 4,2 % par rapport à la prévision actualisée pour 2023 et de 8,8 % par rapport à la réalisation de 2022. Il n’en reste pas moins

la garde à domicile et l’accompagnement des enfants, ou encore l’assistance à domicile et l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques. Resteront également éligibles les activités d’entretien de la maison, petits travaux de jardinage et travaux ménagers, ainsi que les activités de coordination et de délivrance des services proposées par des organismes déclarés, agréés ou autorisés. Les autres prestations pourront continuer d’ouvrir droit au crédit d’impôt, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale : allocations aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés ou encore prime d’activité. En En revanche, certaines prestations de confort, telles que la maintenance, l’entretien ou la vigilance temporaire des résidences principales et secondaires, seront totalement exclues du dispositif. Veuillez conclure. Ces dispositions entreraient en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025. Quel

Selon Clément Carbonnier et Nathalie Morel, il s’agit d’un crédit d’impôt fortement antiredistributif. Plus de la moitié des services consommés concernent des prestations de confort concentrées sur les ménages les plus aisés. Surtout,

des hausses de plafond successives, qui ont eu un fort effet d’aubaine, comme cela est documenté. Nous suggérons donc d’abaisser à 2 000 euros le plafond du montant pouvant être défiscalisé pour les prestations dites de confort. En revanche, nous entendons conserver les plafonds pour les services à domicile liés à l’assistance des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des autres personnes qui ont besoin

« Réduire le coût du crédit d’impôt pour les activités de la vie quotidienne ne relevant pas des politiques en faveur de l’autonomie et de la garde d’enfants. » L’ensemble des économies dégagées par la réduction des services notamment être fléchées pour couvrir les services essentiels, qui souffrent d’un sous financement chronique, ou pour financer le passage de la réduction d’impôt au crédit d’impôt au titre des frais d’hébergement pour les personnes accueillies en Ehpad.

suis aussi le rapporteur spécial de la mission « Remboursements et dégrèvements » que je reprends cet amendement intéressant de Mme Christine Pirès Beaune, mon homologue à l’Assemblée nationale.

quel mot compliqué ! – des crédits d’impôt, notamment en faveur de l’aide à domicile, a accru la dynamique et les coûts de trésorerie pour l’État, qui devraient augmenter de 49 % pour atteindre 2,4 milliards d’euros.

la nature des organismes ni sur la personne morale ou physique qui effectue la prestation. En demandant ces éléments dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts, nous serons à même d’évaluer ce crédit d’impôt, essuie le feu des critiques de différentes institutions. La Cour des comptes constate qu’il ne répond pas aux objectifs qui lui sont assignés et le Conseil des prélèvements obligatoires note à son propos : « Le choix de recourir à un crédit d’impôt avec avance immédiate revient à rapprocher la dépense fiscale d’une logique de dépenses budgétaires sans présenter les mêmes avantages en termes de contrôle. »

dont vont devoir s’acquitter les particuliers employeurs.

à Mme Corinne Narassiguin. Il s’agit de rendre déductibles des impôts les cotisations aux assurances de base à la Caisse des Français de l’étranger pour les cotisants et leurs ayants droit, étant entendu que ces personnes n’ont pas accès au régime de sécurité sociale en France. Quel

de poursuites judiciaires. Non seulement cette situation est inacceptable du point de vue du droit, mais le fait qu’elle provienne d’associations parfaitement connues et bénéficiant de l’aide financière des pouvoirs publics l’est davantage

ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ». En outre, il tend à interdire à ces mêmes associations de fournir des reçus fiscaux, nécessaires pour que les contribuables bénéficient de la réduction d’impôt.

l’avis du Gouvernement

sont des vecteurs essentiels de la cohésion sociale. Ils permettent de tisser un réseau de solidarités locales en proposant des réponses concrètes aux défis du quotidien : isolement, précarité, difficulté d’accès à la culture… culture… Le budget présenté au travers du PLF pour 2025 pourrait, selon France Tiers Lieux, signer la fin de cette politique à destination des territoires. La coupe budgétaire prévue réduirait à néant les efforts pour accompagner ceux qui innovent

M. André Guiol. Cela n’est un secret pour personne : le secteur associatif accuse un manque criant de bénévoles.

et juin 2023. Devant cette situation, il nous faut actionner davantage de leviers pour entretenir et faire grossir notre vivier de bénévoles. Pour rappel, 90 % des associations fonctionnent seulement grâce à ces derniers, selon le réseau associatif Recherches et solidarités. Dans cet esprit, cet amendement vise à démocratiser l’engagement associatif en réduisant les barrières monétaires qui peuvent dissuader les Français les plus modestes de sauter le pas. En effet, la mesure que nous proposons tend à substituer un crédit d’impôt à la réduction d’impôt actuelle afin de rétablir une forme d’équité fiscale et d’égalité entre les bénévoles assujettis à l’impôt sur le revenu et ceux qui ne le sont pas. Les trois

l’implication des 45 000 volontaires qui ont activement contribué à la réussite de cet événement historique. Or il est important de rappeler que les associations et leurs bénévoles jouent au quotidien un rôle fondamental dans notre pays en soutenant des projets au service de la justice sociale, de la solidarité et de la protection des plus fragiles ou en contribuant à la vie culturelle, civique et sportive dans les territoires.

En 2023, les Restos du Cœur ont accompagné 128 000 enfants de moins de 3 ans pour leur assurer nourriture et produits d’hygiène. Le rôle des bénévoles dans toutes ces associations n’est plus à souligner. Toutefois, ceux

? Oui, monsieur le président.

En 2021, dans notre pays, les femmes ont été victimes d’au moins 210 000 viols ou tentatives de viol, soit une agression toutes les deux minutes trente. En moyenne, chaque année sur la période 2011 2018, 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré avoir été victimes de violences physiques physiques ou sexuelles de la part d’un conjoint – concubin, pacsé, petit ami – ou d’un ex conjoint. Parmi ces victimes, 29 % sont âgées de 18 à 29 ans.

d’impôt, dite Coluche, de 75 % pour les dons faits à des organismes d’aide aux personnes en difficulté, dans la limite d’un plafond de 1 000 euros. En 2020, face à l’urgence sociale provoquée par la crise sanitaire, le plafond

Les dons concernés ont ainsi progressé de manière significative, passant de 442 millions d’euros en 2019 à 711 millions d’euros Cette dynamique est vitale pour les organismes comme les Restos du Cœur, la Croix Rouge, les banques alimentaires ou encore le Secours populaire. Ces structures jouent un rôle indispensable dans notre société en venant en aide à celles et ceux qui, chaque jour, peinent à subvenir à leurs besoins essentiels. Dans un contexte marqué par une augmentation du nombre de bénéficiaires, leurs besoins ne cessent de croître. C’est pourquoi il serait bon de maintenir ce dispositif.

au profit des organismes listés à l’article 200 du code général des impôts. Tel est le sens de cet amendement. Le dispositif, ainsi modifié, permet d’allier solidarité nationale et équité fiscale.

le régime permet déjà, sous conditions, aux contribuables non résidents de France, mais résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, de bénéficier des réductions d’impôt, en particulier dans

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de 66 % les dons faits aux organismes, fondations ou associations ayant pour objet la contribution au financement d’un établissement scolaire privé sous contrat ou hors contrat.

Notre amendement fait appel au bon sens paysan : avant de jeter, on répare. Il vise donc à promouvoir l’économie circulaire et la réparabilité des objets, avec la création d’un crédit d’impôt,

je le sais, il y a trop de gens aisés. […] Mais ce n’est pas par une politique qui accentue les prélèvements sur les hauts revenus que vous répondrez au problème difficile du consentement à l’impôt, déjà mentionné. Prélever plus sur les plus hauts revenus ne changera rien si l’on ne change pas le système fiscal. » Il a dit ça

haut niveau de prélèvements obligatoires et taxes de toutes sortes. Pour le moins, le dispositif proposé devrait être borné dans le temps.

permises par l’insuffisante régulation de la captation des ressources publiques par de grands groupes privés, qui privilégient la rentabilité au détriment du bien être des enfants. Parmi certaines pratiques répandues, l’instrumentalisation et l’optimisation de dispositifs fiscaux tels que le crédit d’impôt famille, le fameux Cifam. Dans son rapport de janvier 2024 sur les modèles de financement et la qualité d’accueil des microcrèches, les multiples limites du Cifam. Elle a constaté que ce dispositif avait contribué à l’accroissement des inégalités, parce qu’il bénéficie en majorité aux grandes entreprises, mais surtout parce qu’aucune limite n’a été posée quant au prix unitaire du berceau, lequel a subi de ce fait un fort effet inflationniste. La liberté accordée aux microcrèches en matière de pratiques commerciales a ainsi permis aux grands groupes privés de crèches de pratiquer des tarifs anormalement élevés sur le prix des places, en ciblant principalement les grandes entreprises. Les écologistes rappellent qu’il faut urgemment envisager le redéploiement partiel des moyens alloués au Cifam, source d’inégalités importantes, vers le financement d’un véritable service public de la petite enfance.

en fixant notamment un montant maximal par enfant accueilli. Or le crédit d’impôt est plus large que le seul financement des places en crèche : il concerne également les dépenses de formation, les subventions pour garde d’enfants, etc. Au delà des enjeux rédactionnels,

ne sont pas comprises dans la liste concernée par le II de l’article 1378 du code général des impôts. Notre amendement vise à corriger cet oubli,

Un certain nombre d’infractions sont visées par le code général des impôts. L’amendement a pour objet d’étendre la liste de ces infractions, notamment aux infractions subies par les agriculteurs dans leurs propriétés, en particulier

les dons, legs ou versements effectués au profit de l’organisme condamné ne peuvent plus donner lieu au bénéfice d’un quelconque avantage fiscal. Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à ajouter la condamnation pour délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse aux infractions énumérées à l’article 1378 du code général des impôts. Il s’agit de refuser que les organisations entravant la liberté constitutionnellement garantie des femmes à interrompre leur grossesse puissent obtenir des avantages fiscaux, donc être indirectement financées par les contribuables. Quel est l’avis de la commission ? Je sollicite

l’amendement n° I 1009, qui tend à ajouter la condamnation pour délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse

Le scrutin est ouvert.

pour détailler les modalités d’application de ce texte, prévoit que, dans certains cas, il sera tenu compte non pas de la date effective d’encaissement, mais d’un événement juridique créateur de droits antérieur à cette date. Or les premiers actes de poursuite aux fins de recouvrement interviennent très rapidement après la procédure de contrôle. Dans la pratique, lorsque l’époux solidaire n’a pas forcément encore pris conscience de l’implication, voire de l’existence de la solidarité et qu’il n’a donc pas encore sollicité la séparation

t elle considérablement de l’intention initiale de la loi. Le présent amendement vise donc à préciser l’intention du législateur. La loi du 31 mai 2024, qui vise à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, a introduit une extension du dispositif de décharge de responsabilité solidaire. est notamment prévu que celle ci peut donner lieu à la restitution de sommes déjà recouvrées par le fisc après l’événement attestant de la séparation. que les montants potentiellement restitués soient les sommes « effectivement encaissées » et non les sommes « recouvrées ». Je sollicite l’avis du Gouvernement sur ce point, pour qu’il nous informe des conséquences d’un tel changement sur un texte que nous avons adopté très récemment.

des pourboires de l’imposition sur le revenu et des cotisations sociales pour les années 2025 et 2026. L’exonération des pourboires des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu a prouvé son efficacité depuis sa mise en place, en 2022. En trois ans, elle a permis et aux entreprises du secteur de l’hôtellerie restauration de gagner en attractivité, ce qui crucial dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, et aux salariés de bénéficier d’une reconnaissance accrue de leurs revenus, notamment pour des démarches comme l’accès au crédit. Le dispositif de cet amendement, élaboré en concertation avec la CPME et défendu initialement par la députée Olivia Grégoire, vise à prolonger cette exonération jusqu’en 2026. C’est une mesure de justice sociale, qui améliore les conditions de travail des salariés tout en soutenant un secteur clé de l’économie française et

Cette mesure, vous vous en souvenez, permet aux salariés qui souhaitent augmenter leur activité de convertir en rémunération, avec l’accord de leur employeur, leurs demi journées ou journées de

est à Mme Sabine Drexler. Le Président de la République a annoncé, le 15 septembre 2023, le lancement d’une collecte nationale de dons pour financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants en métropole, et de moins de 20 000 habitants en outre mer. Ces édifices, qui participent à l’identité et au charme de nos villages, sont aujourd’hui en péril : le manque d’entretien et les budgets contraints des communes qui en ont la charge plongent progressivement bon nombre de nos églises, temples et synagogues dans un état de délitement. Afin d’inciter les particuliers à concourir à cette collecte nationale, l’article 30 de la loi de finances pour 2024 porte le taux de la réduction d’impôt de 66 % à 75 % pour les dons effectués entre entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine, dans le cadre de son activité d’intérêt général. Cet amendement tend à élargir le nombre d’organismes collecteurs, au delà de cette seule fondation, à d’autres d’autres fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) qui agissent elles aussi pour la conservation et la restauration du patrimoine, afin que l’ensemble des donateurs bénéficient de manière équitable du même taux de réduction d’impôt.

Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, je ne partage pas

n’est pas acceptable, comme nous en discuterons prochainement. C’est précisément pour cette raison que cet amendement offre une solution plus juste et plus équitable une surtaxe ciblée sur les foyers les plus aisés, qui disposent des capacités contributives nécessaires. Cela a été rappelé : seuls 80 % des foyers étaient initialement concernés par la suppression voulue en 2017.

puis scrutin public solennel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont le